Séance est reprise bonsoir, chers collègue, Madame la Ministre, l'ordre du jour appelle le débat sur quel bilan pour Parcoursup demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, je vous rappelle que dans le cadre de ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur ou oratrice pour une durée de 2 minutes l'orateur disposera alors à son tour d'droit de répartis pour une minute. Madame la Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez répondre après chaque orateur à votre choix vous signalerai, une fois que celui-ci, on a retrouvé une place dans l'hémicycle, la parole et tout d'abord à l'orateur du groupe, qui a demandé ce débat monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons proposé ce débat, non seulement pour dresser un bilan des conséquences de la procédure nationale de préinscription et d'orientation des candidats dénommée Parcoursup, mais aussi pour échanger sur l'université et encore plus généralement sur les missions du service public de l'enseignement supérieur, nos sociétés par leur système productif reste grandement dépendante des matières fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz sur lesquelles elles ont bâti leur essor à la fin du XVIIIe siècle, nul ne conteste plus que les rejets massifs de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont provoqué un réchauffement climatique qui menace aujourd'hui notre existence même, il a fallu près de 3 siècles pour développer une économie exploitant à l'extrême les capacités des énergies fossiles, il ne nous reste plus que quelques décennies pour les abandonner et refonder l'essentiel nos productions sur d'autres ressources, jamais depuis l'aube de l'humanité, nos sociétés n'ont été confrontés à des Dauphy aussi considérable, soyons persuadés que seul le savoir, la recherche et la mobilisation de toutes les intelligences nous permettront de surmonter ces épreuves l'université parce qu'elle forme les esprits dont nous aurons besoin et parce qu'elles participent directement à ce grand effort de surcroît de connaissance devrait être au coeur de nos politiques et un des objets essentiels de nos priorités publiques, or les moyens que l'État lui consacrent ne cesse de baisser proportionnellement au nombre d'étudiants qu'elle accueille bon nombre d'établissements sont au bord de la banqueroute et ne savent pas aujourd'hui comment ils se chaufferont cet hiver, comment expliquer ce paradoxe : comment comprendre cette contradiction entre nous énormes besoins en matière de formation et de recherche et la pauvreté des moyens de l'université, quelle est la cause de ce mal français, il procède principalement à mon avis, du fait que les élites françaises ignorent l'université et parfois la méprise, elle considère de façon générale, qui n'est point besoin de trop investir dans l'université, tant que les grandes écoles continueront d'assurer leur reproduction cette dichotomie entre des grandes écoles bien dotées des universités nécessiteuses est ancienne trouve sans doute son origine dans les réformes napoléonienne, rappelons que l'État octroie aujourd'hui 4 fois plus de financement à un élève de classe préparatoire qu'un étudiant de licence, il n'est pas possible de dresser un bilan de l'orientation et de Parcoursup sans souligner les disproportions de moyens accordés à ces 2 systèmes au sein même du service public par le passé à plusieurs reprises des gouvernements tentèrent de réduire cette fracture, l'intégration des classes préparatoires au sein des universités fut ainsi l'une des mesures proposée par Edgar Faure dans son projet de réforme de l'université, une réaction corporatiste, relayé par des ministres importants de son gouvernement eux-mêmes issus des grandes écoles l'obligea à y renoncer, dans ses mémoires, le général de Gaulle, commenta ainsi cet échec, je le cite, ayant moi-même élargi à l'extrême l'enseignement public je donc à y faire s'instaurer depuis le bas jusqu'en haut, l'orientation et la sélection, il me fut une fois de plus démontré qu'à moins de faire table rase par la dictature ou par la révolution, aucune institution ne peut vraiment être réformée si ses membres n'y consent pas, je cite à dessein, le général de Gaulle car c'est sous son gouvernement que le processus de démocratisation de l'université a connu son évolution la plus radicale entre 1958 et 1968 le nombre de bacheliers généraux se multiplier par trois comme les effectifs d'étudiants qui passèrent de 170000 à 500000 et celui des ingénieurs qui doubla je rappelle que le CNRS compter 6000 agents en 1958 et 16000 en 1968 cet accroissement sans équivalent fut pensé et organisé pour accompagner des investissements massifs dans tous les domaines de la science et de la technologie, il fallait des cerveaux pour les programmes très ambitieux, consacré notamment aux industries nucléaires et spatiales Maurice Duverger, a résumé cette politique par cette formule dans les sociétés industrielles le malthusianisme universitaire est une absurdité, alors que nous sommes présentement confrontée à des objectifs technologiques bien plus considérables cet exemple d'une planification réussie qui lie l'augmentation de l'offre de formation à l'accroissement des moyens de la recherche doit être pris pour exemple, il est inconséquent de vouloir porter l'effort de recherche et développement de la France à 3 % de son PIB, sans investir massivement dans ses universités, la difficulté, je le conçois et d'organiser cet effort de formation pour qu'ils participent au développement de nos capacités de recherche tout en préservant la nécessaire autonomie pédagogique des universités et sans amoindrir amoindrir les ressources d'une recherche fondamentale dont les apports ne seront effectives que dans plusieurs décennies cette équation très difficile à résoudre oblige préalablement l'État à réfléchir à une programmation à la discuter avec les scientifiques et à faire une fille et des choix politiques autant de perspectives singulièrement ignorés par la mal nommée loi de programmation de la recherche, pour être plus concret, j'aimerais prendre l'exemple de la formation des médecins pour réduire les dépenses de santé, il a été décidé il y a plusieurs dizaines d'années, de diminuer le nombre de médecins formés, la réussite de cette politique est telle qu'il faut maintenant renverser la logique pour réduire la carence de médecins si chaque université organise en totale économie son recrutement, il est douteux que la somme des choix de ces établissements fasse une politique nationale dans son rapport sur la mise en oeuvre des réformes de santé notre collègue la sénatrice Sonia de la Provoté a proposé que le recrutement des étudiants en médecine obéissent à des objectifs infra-régionaux définis nationalement pour tenter de mieux satisfaire les besoins des territoires, la logique qui sous-tend la procédure dite de Parcoursup est radicalement inverse, sa seule finalité et de donner aux établissements les moyens techniques d'ajuster leur recrutement à leurs moyens budgétaires Parcoursup leur permet de gérer la pénurie en conformant les demandes au moyen Parcoursup et le lit de procureur de l'enseignement supérieur, les termes du débat que nous vous proposons dépasse donc la comparaison comptable des mérites respectifs d'APB et de Parcoursup ou la simple revendication de l'abrogation de cette dernière procédure si nous défendons encore le principe d'une université républicaine au service de la nation a prenante si nous voulons toujours Rendre la raison populaire comme le souhaitait Condorcet, si nous estimons, de même que l'université peut être un outil efficace de l'aménagement du territoire et de la satisfaction d'objectifs scientifiques à long terme, alors il convient de réfléchir ardemment aux conditions d'un dialogue renouvelé entre l'État garant d'une planification ambitieuse et les universités qui la mettent en oeuvre dans le respect de l'autonomie des équipes pédagogiques, je vous remercie.

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias tout d'abord, je dois vous reconnaître au groupe CRCE et à vous-même, monsieur Pierre, Un sens aigu du timing pour Parcoursup en tout cas, puisqu'effectivement, ce matin même à sept ouverte la phase dite de paramétrage des formations qui ouvrent en quelque sorte cette cession Parcoursup 2023, il est donc à point nommé, mais avant de revenir sur Parcoursup, quelques mots peut-être à votre en réponse à votre intervention, d'abord je voudrais vous dire que je vous rejoins sur le fait que l'université avec un grand tu doit être au coeur de nos politiques, alors vous imaginez que ma réponse demanderait plus de 2 minutes, mais je voudrais vous en dire quelques mots, oui, nous défendons encore et toujours le principe d'une université républicaine d'un service public qui doit revoir cette notion de méritocratie, mais à l'aube du XXIe siècle, oui, nous avons toujours les mêmes missions coeur de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche mais inscrite dans notre époque notre société et tous les défis que vous avez cités que nous avons à relever aujourd'hui et demain, c'est pourquoi avec conviction et en toute responsabilité, nous allons effectivement mettre en place ce dialogue renouvelé avec les universités, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de l'ESR au niveau de Parcoursup rapidement, il faut rappeler au moment de ce débat que la procédure Parcoursup assure un échange entre les lycéens et les enseignants des formations post-bac, que la loi du 8 décembre 2018 a effectivement organiser ce débat qui nous réunit, ce soir, et l'occasion, je n'en doute, vraiment pas de revenir sur le chemin parcouru depuis 5 ans au service de plus des 4 5 millions d'usagers qui ont utilisé Parcoursup depuis 2018 et de discuter des axes qui nous permettront de continuer ce travail de constantes améliorations dont Parcoursup a encore besoin aujourd'hui, j'en suis pleinement consciente et je voulais vous le dire dès le début, je vous remercie. Merci madame la ministre, dans la suite du débat, la parole est à monsieur Thomas Dossus du pour le groupe Écologie solidarité et territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, et je tiens tout d'abord à remercier le groupe communiste pour l'inscription de ce débat essentiel à notre de notre il y a beaucoup de choses à dire sur le système dont nous faisons le bilan aujourd'hui, celui de Parcoursup, créé par la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants de mars 2018 Parcoursup a organisé le système d'admission dans les formations d'enseignement supérieur pour la 4ème année c'est la 4ème rentrée cette année, destiné à remplacer le système d'admission post-bac post-bac APB, le nouveau système se voulait plus efficace et plus juste, celles et ceux qui en parlent le mieux sont les étudiantes et les étudiants et élite l'étude Ipsos-réalisés chaque année sur plus de 1000 néo-bacheliers à ce sujet, permet d'avoir un aperçu de l'expérience utilisateur pour reprendre les termes de la Start-Up, nation, les résultats sont sans appel : si 74 % des interrogés trouver le système fiable en 2020 il n'étaient plus que 66 en 2021 et 57 en 2022, c'est la même chose et même pire pour l'équité du système 48 % estimaient que Parcoursup était juste en 2020, ils ne sont plus que 28 % en 2022, idem pour la transparence 60 % en 2020 48 % en 2022. Et le seul indicateur en constante augmentation et celui du stress généré par les pour les futurs étudiants 77 % était stressé par le le système en 2020 contre 83 % en 2022, en résumé, pour les lycéens aujourd'hui Parcoursup ni fiable ni juste ni transparent, à peine la moitié trouve qui lui permet d'exprimer ses besoins et 8 lycéens sur 10 le vivent comme un stress alors on entend souvent dire que par Parcoursup est perfectible, mais ces chiffres nous indique plutôt que tout est à revoir, d'autant que les derniers répondant sont les premiers qui ont vécu tout la coupe tout le lycée de la seconde à la terminale, avec ce système, pour comprendre les raisons du rejet grandissant souvent le capot et reprenons pas point par point les 2 objectifs que s'étaient fixés les inspirateurs de ce système, efficacité et justice en d'autres termes parcoursup permettent efficacement, de construire un parcours d'étude choisi pour un ou une bachelière concernant l'efficacité, cette notion est plus que discutable, là où le système qui était plutôt médiocre d'APB proposait une hiérarchisation de 24 choix de filières pour les futurs étudiants avec 3 phases admission à date fixe et un algorithme assez obscur Parcoursup ne permet que 10 choix par candidats qui seront depuis cette année seulement hiérarchisée, avec des réponses qui peuvent intervenir à tout moment et demande la confirmation en moins de 5 jours une sélection avec des algorithmes locaux différents selon les UFR, le tout est organisé en plusieurs phases, une principale une complémentaire, une saisine possible une commission ad-hoc pour les restant à la fin du Provisy et prévisible pour une bonne partie des étudiants, les choix sont souvent faits par défaut, anticipant des critères de sélection flou ou opaques et mal accompagné, auxquels s'ajoutent des délais d'attente parfois impossible qui engendre un stress permanent. Au terme de la première phase de sélection mi-juillet environ 10 % des candidats, soit plus de 90000 personnes se retrouvent toujours sans affectation. Sur la justice du du système ensuite qui est à mon sens véritablement le coeur du problème parcoursup les chaque UFR établir ces critères qui ter qui on pouvait en douter sans douter pardon sont basés principalement sur les notes, mais aussi sur les lycées d'origine ou encore sur les j'outils automatisés d'aide à la décision pour ne pas dire d'aide à la sélection, la Cour des comptes a décrit, je cite un fonctionnement nébuleux des commissions d'examen des voeux et des critères de plus en plus automatisés et demande de rendre publiques des algorithmes utilisés par ces commissions pour l'ensemble des formations, il y aurait beaucoup à dire, notamment sur l'incapacité de Parcoursup à combler les manques des services administratifs en sous-effectif chronique depuis des années sur le poids qui pèse en terme horaire sur les équipes éducatives qui doivent s'occuper maintenant des procédures de classement sur le marchepied que constitue la plateforme pour les formations privées sur le coût exorbitant du dispositif aux seuls attendu le départ, efficacité et justice, on peut dire, on peut déjà conclure à un double échec, madame le ministre, il est temps d'écouter les futurs étudiants, le système actuel est un système de tri souvent arbitraire qui ferme un certain nombre de parcours et de filières à de très nombreux étudiants et ouvrent grand les portes des filières privées au delà d'une réforme en profondeur des procédures d'admission et de l'enseignement supérieur, ouvrons et investissons ouvrons de nouvelles filières en adéquation avec les aspirations grandissant des étudiants pour le savoir du monde de demain investissons massivement dans l'autre université notre recherche publique en développement, les campus en créant de nouvelles unités de formation pour accueillir les bacheliers dans les filières qui le souhaitent et non pas dans les filières, par défaut, l'université de demain est un un idéal qui doit préfigurer la société de demain inclusive égalitaire, solidaire Parcoursup ne contribue pas à nous mener vers cette université au service de l'émancipation, il nous en écarte, c'est pourquoi il est temps de le repenser de fond en comble, je vous remercie. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, donc bien entendu croyez monsieur le sénateur. Vous êtes contre, vous l'avez dit, vous vous êtes contre, et vous êtes même contre le fait de garder Parcoursup et moi aujourd'hui, je suis pour l'améliorer pour continuer à améliorer une plateforme qui existe depuis 5 ans, où nous avons un retour d'expérience depuis 5 ans, plutôt que de mettre à nouveau une nouvelle plateforme pour accompagner nos étudiants vers la réussite, vous avez cité des chiffres effectivement il y a eu ce ce ce ce rapport. Sauf que nous avons chaque année où vous pouvez comparer les chips, je voudrais vous en citer aussi qui sortent du même rapport l'évolution de ces chiffres est plutôt positif, partout où vous regardez en grande majorité au cours de ces années une Lingemann majorité des lycéens aujourd'hui apprécient le fait de retrouver sur Parcoursup toutes les formations reconnues par l'État 89 % % c'est vraiment un outil de vitrines de nos formations accessibles pour tous, de tous les étudiants et de toute la France et la liberté de formuler leurs voeux quatre-vingt-six % les indicateurs liés à la phase d'admission progresse également 72 % sont satisfaits des réponses, des formations à leurs voeux, c'est plus de points par rapport à 2021 et 68 % sont satisfaits des délais de réponses 4 points par rapport à 2021 aujourd'hui ces délais, pour la première propositions sont liées sont au bout de quatre de jours pour les étudiants, alors oui et j'en suis consciente, je vous l'ai dit, il y a des améliorations à faire, et avec mon collègue PAP Ndaye nous allons-y travailler pour l'orientation pour améliorer l'argumentation pour diminuer ce ressenti de stress maîtresse qui est quelque part lié à l'avenir de, de, de ces jeunes, donc une partie du stress, je dirais normale et une autre sur lequel nous devons agir je voudrais vous dire que, aujourd'hui, les dix feux sont faits pour les étudiants sans hiérarchie des voeux afin que l'étudiant jusqu'au bout et le choix de la formation qui lui ont proposé, alors qu'à APB vous choisissiez hein dit veut en février et vous aviez le 9ème veut sans savoir si votre dixième été pris en juin, en juin, juillet, aujourd'hui c'est une amélioration qui place l'étudiant au centre et ce système, ce n'est pas un système d'algorithmes, c'est un système de choix où l'humain est au centre, puisque ces comités d'examen sont avec des enseignants, des enseignants du supérieur en lien avec les lycées et qui sont là, je peux vous le dire, pour avoir pendant 30 ans était à leurs côtés, être là pour le bien de nos élèves le bien de nos étudiants et nous allons-y travailler avec eux. Merci Merci madame la ministre, je, je sais que nous apprécions que vous répondiez systématiquement, je vous demande juste d'être vigilante sur les deux minutes pour que tout le monde puisse voilà mais on on apprécie d'avoir une Ministre qui répondent, c'est pas toujours le cas. Non, non, je ne donnerai pas de nom, la parole est à madame Nicole Duranton pour le groupe des pays. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, quel bilan pour Parcoursup retour d'expérience depuis sa création en 2018 la plateforme fonctionne de mieux en mieux comme vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, crée Parcoursup créé par la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, c'est en effet un système qui peut être encore améliorée grâce au retour d'expérience, mais dont les carences ont néanmoins été corrigé par le ministère, chaque année, il est impossible d'obtenir un résultat parfait dès les premières années, mais le gouvernement a su garder une oreille attentive et prendre en compte les demandes des utilisateurs, comme vous le savez, les lycéens ou étudiants en recherche d'une réorientation y compris sous statut apprentis ont ainsi accès à plus de 21000 formation supérieure, dont plus de 7000 en apprentissage, si la phase d'information officielle ouvrira pour cette année, le 20 décembre les jeunes peuvent d'ores et déjà, comme vous l'avez indiqué se connecter à la plateforme pour y découvrir les formations, cette première phase de novembre avant le conseil de classe est essentielle pour que chacun puisse préciser l'idée qu'il fait de son futur cette information constitue le 1er degré, de l'égalité des chances, les établissements sont encore en train de calibrer leur présentation en 2022, la plateforme a connu 936000 candidats, dont 622000 lycéens, on a pu entendre que Parcoursup ne leur laisse pas assez de choix 11 6 millions de voeux et sous-voeux ont été formés pour des formations en statut étudiant, soit plus de 12 veut en moyenne par élève, on a pu entendre que Parcoursup n'accompagnait pas tous les jeunes et que certains étaient laissés pour compte, pourtant à l'issue de la phase principale les candidats sans proposition peuvent solliciter l'accompagnement des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui conseille les recteurs, on a pu entendre que Parcoursup était trop opaque, or les jurys doivent désormais produire un rapport public sur les critères ayant motivé les décisions d'admission mais surtout de non-admission des lycéens, on a pu entendre encore que Parcoursup ne compensait pas suffisamment les inégalités structurelles entre les catégories socio-professionnelles et les territoires, notamment dans la ruralité, en effet, comme le rappelle la Fédération des territoires aux grandes écoles, qui agit directement auprès des lycéens, les territoires ruraux 17 % des lycéens généraux et technologiques fournissent à eux la seule moitié, seule seule la moitié des effectifs des grandes écoles, les élèves parisiens ont 3 fois plus de chances d'accéder aux études qu'ils appellent de leurs voeux, c'est une réalité et Parcoursup en tentant de valoriser les dossiers et l'expérience personnelle de chacun porte aussi cet objectif, il faut un système national ambitieux comme ce dispositif si l'on veut que l'égalité des chances soit réel que proposent les détracteurs de Parcoursup, en remplacement un système fondé seulement sur les bulletins scolaires qui néglige les parcours individuels, un système linéaire, laissant la main à l'arbitraire, un système de recrutement totalement ouvert où chaque école fait son marché et qui créerait une confusion totale

autant de défauts qui faisait de l'orientation des lycéens, un véritable parcours du combattant et qui a été largement critiqué sur Parcoursup les voeux ne sont plus classés les établissements étudie tous les dossiers reçus et l'étudiant peut se réserver le droit d'attendre une proposition qu'il estime plus intéressantes, le moteur de recherche favorise la mobilité des étudiants et leur capacité de choix, l'abandon du principe de classement des voeux a permis aux boursiers de moins s'autocensurer doit-on regretter les files d'attente devant les unir les universités doit-on regretter le tirage au sort d'APB Parcoursup apporte une réponse efficace à de défauts, mes chers collègues of au front ensemble à améliorer Parcoursup au service de notre jeunesse, au lieu des 2 critiquer ce fameux algorithme alors que ce sont bel et bien des agents qui travaillent derrière cette plateforme. Madame la Ministre, en juillet dernier lors d'une séance de questions d'actualité au gouvernement je vous interroger au sujet des lycéens qui n'avait pas encore reçu de réponse favorable sur Parcoursup, vous m'aviez alors souligné que ce n'était pas qu'un outil, mais aussi un processus humains avec l'accompagnement de tous nos élèves par des milliers d'enseignants et professionnels de l'orientation en lycée et dans les rectorats 9 lycéens sur 10 avaient alors reçu au moins une proposition vous aviez très justement affirmé qu'il est bien d'entrer dans l'enseignement supérieur, mais qu'il faut surtout réussir, or en 2 ans entre 2018 et 2020, le taux de réussite en 1er cycle et en licence est passé de 40 à 45 % et le taux des boursiers de 20 à 25 c'est une réussite dont je me félicite ainsi que mon groupe le RDPI cette réussite reste perfectible, mais la procédure a déjà gagné en transparence et en lisibilité en 2022 la phase principale a été accéléré pour améliorer le temps de réponse aux candidats votre projet Madame la Ministre, pour la session 2023 et d'améliorer l'objectivité du processus et sa lisibilité, Madame la Ministre, où en est-on aujourd'hui du développement des améliorations continues prévues sur cette plateforme Parcoursup, qui évolue dans le bon sens, depuis sa création, je vous remercie. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la scène. Nicole Duranton, d'abord merci tout d'abord pour vos propos qui permettent effectivement de resituer les enjeux, les progrès et les améliorations Parcoursup n'est qu'une plateforme c'est vrai, hé bien des responsabilités sont en jeu dans l'accès à cet enseignement supérieur, il ne faut pas le cacher, et c'est pour cela que le travail d'amélioration que vous avez évoquée doit être menée avec toutes les parties prenantes du secondaire et du supérieur Parcoursup a fait des progrès et engager des améliorations pour mieux servir d'abord les intérêts des jeunes et écouter les étudiants, nous le faisons depuis 5 ans et les lycéens dans l'étude d'opinion publiée en septembre, en témoignent aussi, oui madame, madame la sénatrice l'accompagnement à l'orientation au lycée existe et nous allons continuer à l'améliorer, oui parcoursup apporte des informations pour faire son choix et, là aussi, dès cette année des progrès arrive, oui, les délais de réponse se sont améliorés et nous allons diminuer ces délais, ainsi que la transparence des critères pour Parcoursup je voudrais vous dire aussi que cette année, il ne restait que 160 étudiants après après les CAES plus que 33 après les avoir suivi un par un pour leur intégration dans l'enseignement supérieur, nous nous engageons donc à continuer ses améliorations sur toute tous ses volets, dès 2023 et sur les 4 axes ce trajet stratégique que je vous présenterez. Merci. Parole maintenant à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tenter de tirer un bilan constructif de Parcoursup conduit à éviter 2 écueils, un optimisme débridé devant la capacité de l'outil à Paris un nombre important d'étudiants avec de multiples formations sans même questionner la pertinence de cet appariement et à l'inverse, une critique sans mesure qui tend à confondre l'algorithme Parcoursup avec la procédure Parcoursup en somme, éviter tout manichéisme j'aborderai donc ce débat à travers une problématique générale de quoi Parcoursup de par ses sous-jacent ses modalités, ses implications est-il finalement le révélateur en matière d'orientation des jeunes, si nous nous référons à la loi originale de 2018 la création de Parcoursup répondait à un double objectif: mieux orienter et garantir la réussite des étudiants, l'orientation étant la condition sine qua none de cette réussite, or en l'état, je crois que Parcoursup révèlent la prédominance d'une conception de l'orientation, celle de l'appariement, celle de la gestion urgente des flux étant donné la démographie estudiantine conséquence directe: les étudiants non plus nécessairement le choix de leur orientation, ils peuvent d'ailleurs parfois le subir en particulier lorsqu'il se destine aux filières en tension, leur liberté de choix devient alors conditionnel et c'est une réalité que notre groupe n'a eu, ne cesse de dénoncer, qui va à rebours de ce creux préconisait le Césaire dans son rapport de 2018 sur l'orientation des jeunes, il n'est pas admissible que le manque de places dans certaines formations contraignent les étudiants à accepter des choix parfois éloignés de leurs voeux 1er malheureusement et mécaniquement, cette tendance est aussi de plus en plus prégnante à l'entrée en master ainsi Parcoursup révèle l'institutionnalisation d'une sélection partielle à l'entrée dans le supérieur pour endiguer la pénurie de places résultant du manque de moyens pour la justifier, certains ont avancé qu'il valait mieux cette sélection que l'échec qui prévalait en licence, auparavant, je répondrai que ni la généralisation de l'échec ni la généralisation de la sélection ne sont souhaitables et s'il était insatisfaisant de se reposer uniquement sur le principe d'égal accès au supérieur sans oeuvrer concrètement à la réussite de chaque étudiant, il est tout aussi inacceptable de fermer a priori certaines portes de certaines filières, censé être ouverte à tous et toutes, dès lors que la sélection est de mise, l'enjeu de son acceptabilité par les candidats devient centrale, c'est pourquoi l'évolution vers le système Parcoursup a entraîner des modifications des transformations parfois positive dans les modalités d'orientation des jeunes,

en termes d'orientation, les améliorations sont de 2 ordres : en amont, il y a une vraie amélioration d'information mais vous l'avez dit, Madame la Ministre, mise à disposition des candidats Parcoursup est un portail parfois vertigineux d'ailleurs qui comprend des attendus nationaux, locaux pour chaque formation leur taux d'insertion professionnelle et cependant, il convient de ne pas omettre que rendre accessible information ne signifie aucunement qu'elle sera décrypté comme il se doit, d'où l'importance, une fois de plus, de l'accompagnement dans l'orientation et on avale le début n'accompagne d'un accompagnement personnalisé en licence avec ou ici, sur ce point madame la Ministre, il serait opportun d'avoir une évaluation nationale sur la mise en oeuvre dès ou ici dans les établissements du supérieur pour analyser les freins ainsi que peut-être les aménagements auxquels procéder pour rentre le dispositif plus opérant, rappelons que le législateur et singulièrement au Sénat vous rappeler, mes chers collègues, a concédé la création de Parcoursup sous réserve de l'effectivité de ces modules complémentaires devant permettre aux étudiants de se mettre à niveau poursuivent l'orientation de leur choix, pour ma part, je pense que cet accompagnement doit être encore plus renforcée, plus personnalisé, car il est la clé de la réussite des étudiants, d'autre part Parcoursup révèle un changement profond en matière de responsabilité dans le processus d'orientation, d'aucuns d'ailleurs en est voté un transfert de responsabilités d'abord vers les universités, les équipes pédagogiques qui, à travers les commissions d'examen des voeux sont maintenant responsable de la sélection qu'elles peuvent effectuer et elles font un travail, vous l'avez dit ma la c'est vrai très important qu'on peut saluer ce changement de paradigme corollaire de l'autonomisation croissante des universités, explique le combat que nous avons menées en faveur de la transparence des algorithmes locaux combat porté en commun

il est indéniable que la transparence, a progressé de 1000 depuis 2018 malgré les dénis refus répétés, je peux le dire de la précédente ministre mais elle peut encore être raffermi sans pour autant porter atteinte au secret des délibérations se transpercent opère aussi envers les étudiants qui sont rendues encore plus responsables de leur orientation de lecture complémentaires, sont possibles à cet endroit, l'une meilleure hâtive obliger les étudiants à penser leur projet d'orientation plutôt au lycée ah le formaliser, de manière plus détaillée explicite et positive, cela les rend encore plus acteurs de leur orientation les conduit à se l'approprier et facilite la transition vers le supérieur, je pense notamment au projet de formation motivés ou même à l'affiche à venir, l'autre plus nuancée, dès lors que nous raisonnons concrètement dans le monde de Parcoursup tout se passe comme si les étudiants étaient égaux devant l'orientation, or les sociologues de l'éducation, l'ont démontré depuis longtemps en l'espèce comme dans dans dans nombre de domaines égalité réelle ne prévaut et d'ailleurs la mission d'évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur de 2020 réalisés par l'Assemblée nationale ne s'y trompe pas, si l'octroi d'un second professeur principal notamment dédié à l'orientation, la consécration de deux semaines destiné à l'orientation en terminale et la mise en réserve de 54 heures sur l'ensemble du lycée sont bénéfiques, leur application et leur contenu sont parfois très inégaux et très aléatoire, pire, beaucoup de professeurs principaux ne cesse, tu ne s'estiment pas suffisamment formés, si bien que plusieurs académies ont fait part de leur dit. Difficultés de recrutement, beaucoup de chefs d'établissement aussi pense devoir être formée à l'orientation ces statistiques. Explique pourquoi près d'un tiers des lycéens n'ont parfois pas bénéficier de conseils au moment de leur choix d'orientation dans ce contexte, il est plus aisé de comprendre le sentiment d'injustice et d'amertume qui peut saisir les étudiants lorsqu'ils sont refusés dans la formation de leur choix, parce que finalement, il se retrouve responsable d'un échec qui n'est pourtant pas le leur, naturellement Parcoursup n'est pas la seule cause de ce déficit dans l'accompagnement dans l'orientation des élèves, c'est la raison pour laquelle on introduction, souvenez-vous, j'ai plutôt évoquer Parcoursup comme un révélateur, peut-être plus que toute autre considération Parcoursup révèle finalement le lourd investissement qu'il reste à réaliser pour structurer et à améliorer encore notre politique d'orientation qui a constitué depuis des décennies un talon d'Achille de nos politiques publiques car la politique d'orientation et le viatique par lequel lutter efficacement contre les déterminismes de toute nature et par lequel accroître la mobilité sociale, elle est d'autant plus indispensable que le système de l'enseignement supérieur, se caractérise par une forte étanchéité entre les filières, lesquelles sont héritées de secondaire et par des passerelles, encore trop rares, si la politique d'orientation n'est ni proactive ni correctives ni compensatoires alors les étudiants se retrouvent enfermés dans une trajectoire qui ne peuvent plus maîtriser et la moindre inflexion peut jouer, chers collègues, mais je ne vais pas m'étendre la réforme de l'enseignement des mathématiques au lycée, regardez les conséquences qu'il y a eu très vite et très profonde en réalité l'orientation ne s'arrête pas aux au moins trois, plus trois elle s'avère un processus long, complexe intime parfois lié aux conditions personnelle de chaque élève, le César dans son rapport avait parfaitement intégré cette dimension en préconisant de passer de procédures ponctuel un parcours progressif, ce qui implique tout au long de la scolarité, un travail de déconstruction des déterminismes sociaux et un accompagnement personnalisé de chaque élève pour construire son futur désirable alors en conclusion, je voudrais vous dire que le caractère vital de cet accompagnement et d'autant plus fort que les chercheurs ont mis en Herzberg à quel point dans le secteur de l'éducation, les inégalités ce sédiment de ce cumul atteignant parfois leur paroxysme leur paroxysme au moment de la procédure car Parcoursup matérialiser justement toutes ces inégalités passé et dans certains cas les reproduire, autrement dit Parcoursup pourrait être le produit de notre système scolaire alors l'enjeu est primordial, Madame la Ministre, car elle compte il concerne un investissement massif dans notre politique d'orientation, mais aussi dans l'enseignement supérieur, c'est un enjeu démocratique majeur, je vous remercie. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Sylvie Robert. D'abord, vraiment merci, merci infiniment pour votre intervention qui, pour moi, pose au fond les vrais enjeux de l'accès à l'enseignement supérieur, ou en tout cas parmi certains enjeux que vous avez relevé en particulier sur la politique d'orientation l'accompagnement à l'orientation au centre du dispositif cela du dispositif cela exprimé notre conviction que pour être en tous points démocratique, notre système éducatif devait effectivement faire le choix de donner une vraie visibilité à l'éducation à l'orientation et à l'aide au choix des professeurs principaux, vous l'avez dit, ont été désignés en classe de terminale des ressources ont déjà été développés et cela se voit dans les lycées, comme en témoignent les études d'opinion ou le progrès que nous avons vu jusqu'à présent, mais bien sûr, il faut faire mieux en accompagnant beaucoup de monde, mais effectivement davantage les professeurs principaux en les aidant, en quelque sorte à accompagner leurs s'élève qui s'intéressent à leur formation post-bac post-bac dès les premières années au lycée c'est l'ambition que nous avons que nous donnons avec le ministre de l'Éducation nationale et nous y travaillons, en particulier avec l'Onicep, alors je voudrais aussi revenir, vous avez dit donc sur cet accompagnement, cette orientation, on va y travailler. Je voudrais revenir sur le bilan, Daewoo ici le bilan ici est effectivement quelque chose de de qui sera fait d'importants dans le cadre de ce développement du lien moins trois, plus trois et, oserais-je dire avec un focus particulier sur le plus, hein, à l'entrée de l'université ou dans dans le je voudrais vous dire que 1700 dispositif ou ici aujourd'hui et 2700 étudiants en bénéficier en 2022 mais un une vraie évaluation doit être fait je vous rejoins aussi sur la notion de passerelle aujourd'hui nos étudiants ne peuvent pas avoir un parcours linéaire et un parcours de réussite, c'est un parcours d'accompagnement fait de passerelle d'écoute et de suivi, je vous remercie. Et nous continuerons à travailler dans ce sens et à votre votre analyse merci beaucoup. Merci madame la Ministre, la parole est à notre collègue Céline Brulin pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les résultats de la plateforme Parcoursup sont désolant, le ministère a beau indiquer que seuls 160 lycéens n'ont pas trouvé de place ce sont en fait plusieurs dizaines de milliers de bacheliers qui n'ont pu accéder à l'enseignement supérieur cette année, Parcoursup est un instrument de gestion de la pénurie au sein de l'enseignement supérieur depuis 2008 le budget par étudiant ne cesse de baisser et le taux d'encadrement de régresser entre 2012 et 2017 seuls 19 universités sur 68 ont vu la part des enseignants titulaires augmenter et seulement 12 d'entre elles, leur taux d'encadrement s'améliorer timidement cela à de lourdes conséquences pour toute la société ainsi alors que nous, mais manquons de médecins dans de plus en plus de nos territoires, alors qu'il y a pourtant une véritable affluence des candidatures pour les études de santé sur Parcoursup puisqu'avec les études, enfin avec les instituts en soins infirmiers, ce sont celles qui sont les plus demandés, les capacités d'accueil dans nos universités empêche non seulement des jeunes d'épouser des carrières auquel ils aspirent, mais également de lutter efficacement contre la désertification médicale et la saturation de notre système public d'enseignement supérieur poussent de plus en plus d'élèves à se tourner vers des formations privées 25 % des étudiants du supérieur, ils sont inscrits et rien que pour l'année 2021 2022 le marché privé de l'enseignement supérieur a progressé de 10 quand tu le périmètre de l'université ne le faisait que de 0 4 % Parcoursup est aussi un système qui accroît les inégalités, renforce que la réforme du lycée du bac renforce en faisant peser sur les épaules d'adolescents de 15 16 ans, la responsabilité du choix des disciplines de spécialité afin qu'elles correspondent aux attendus de l'établissement d'enseignement supérieur, qu'il qu'il soit, souhaite intégrer et les 54 heures d'orientation dispensés par les profs principaux sont d'un bien maigre secours face à cela, selon une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, 56 % des étudiants de classes populaires indique que leurs proches ou leurs familles ont permis de construire leur choix d'orientation, ils sont 76 %, dans le cas des classes dominantes, le constat fait par le Conseil d'analyse économique et implacable, un jeune issu d'une famille aisée à 3 fois plus de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un jeune issu d'une famille aux revenus modestes disparités entre jeunes donc disparités aussi entre universités, celle de Paris, hein, voit le nombre de néo-bacheliers avec mention qu'à l'accueil progresser significativement à l'inverse, la part de ceux qui ont plus de 19 ans diminue l'université d'Evry, voit elle diminuer sa part de néo-bacheliers généraux ainsi que ceux avec mention, on pourrait aussi évoquer les bacheliers des filières professionnelles qui accèdent de plus en plus rarement à la licence, avec une baisse notable de ces derniers dans les filières Staps certains diront sans doute que nous avons une lecture idéologique de Parcoursup et de ses algorithmes alors et 11 ans une lecture pragmatique et voyons si la plateforme assure la régulation des métiers dont notre société a besoin, hé bien, pas davantage le récent rapport de notre collègue Catherine Deroche et là, de la commission d'enquête sénatoriale sur la situation de l'hôpital a montré par exemple que les candidats à l'entrée en institut de formation en soins infirmiers étaient près de 690000 en 2021 contre 180000 il y a 4 ans lorsqu'existait le concours de quoi résorber la pénurie de soignants que nous connaissons aujourd'hui, et bien au contraire, on connaît actuellement un taux d'abandon sans précédent durant la formation qui allumant qui alimente la pénurie, la trop faible mixité dans certaines filières, la ségrégation sociale à l'Oeuvres sont en effet un problème qui dépasse largement la seule éthique 2000 bacheliers issus du bac pro bac pro techno ST2S par exemple sciences technologies de la santé et du social, ce qui représente quand même plus de 20 % des effectifs de ce bac se sont retrouvés exclus en 2019 via Parcoursup de la formation d'infirmier à laquelle il s'était pourtant destinée en choisissant précisément ce Baccalauréat, combien d'autres ont connu le même sort, depuis il nous manque aujourd'hui, notamment dans nos hôpitaux, de même pour ce qui concerne les études de médecine nous ne auront pas les déserts médicaux qui gagne nos villes moyennes et nos zones rurales tant que seront quasi exclusivement des jeunes issus des filières scientifiques ayant obtenu leur bac avec mention très bien et grandi dans les métropoles ou les villes universitaires qui y accéderont, la démocratisation de l'enseignement supérieur et donc une nécessité pour répondre aux besoins de notre pays, tout comme l'investissement massif dont il doit faire l'objet. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, mais c'est mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices madame la sénatrice Céline Brulin, alors je ne ferai pas de bataille de chiffres, car vous le savez comme. Pour vous comme pour moi, chaque étudiant est important donc peu importe 60, nous essayons de les gérer un à tous, vous posez la question des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, vaste question, vous comprendrez peut-être que ces inégalités existaient bien avant Parcoursup et je mets même essayer non pas de vous convaincre mais de vous montrer que Parcoursup apporte une contribution à ce défi, aussi, de l'égalité d'accès et de réussite des étudiants ne serait-ce qu'en mettant à disposition de tous les mêmes informations et les mêmes opportunités de faire des voeux librement madame Duranton la rappeler, entre 2018 et 21 le taux des lycéens boursiers admis sur Parcoursup a progressé de 5, de 25 à 25 % grâce au taux de boursiers boursiers volontaristes, voulus par la loi de 2018 et géré par Parcoursup pour 2022, ce sont près de 12300 lycéens boursiers qui ont été admis dans la formation de leur choix et qui n'aurait pu être admis sans les taux de priorité instauré par la loi, Where orientation réussite étudiant il y a des exemples très concrets, l'intégration sur Parcoursup de Sciences Po Paris a permis d'attirer davantage de pour scier on compte parmi les ennemis 12 pour 100 de boursiers du secondaire en 2022 contre 5 % en 2020 et 3 8 des ennemis de 2019 pour lutter contre cette auto-censure, nous avons aussi promu les parcours des élèves en cordées de la réussite auprès des formations, cela a aussi eu des effets tangibles, 6, 7 points de taux de propositions pour les bacheliers professionnels en cordées de la réussite par rapport à ces mêmes lycéens or cordée je fais effectivement, moi aussi, de l'égalité d'accès de réussite des étudiants ma priorité et c'est pour cela que nous avons fait le choix avec Parcoursup de la priorité donnée aux bacheliers technologiques à l'accès au but de la priorité donnée aux actes, aux bacheliers pro pour l'accès au BTS et du soutien de 500 euros à la mobilité des lycéens lycéens boursiers ainsi que du droit aurait examen avec la pluie, du recteur pour les candidats en situation de handicap et je pourrais vous en citer d'autres, et je suis prêt à travailler bien sûr, merci. la parole est maintenant à notre collègue Jean Grey pour le groupe Union centriste. Bien, monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, combien d'entre vous sont des parents ou des grands-parents inquiets devant devant devant le désespoir de leur enfants ou petits-enfants face à la difficulté des choix à faire pour leur avenir, je voudrais partager si le vécu de de jeunes Antoine 20 ans en 2020 à formuler, 9 au total, au 1er soir des réponses, il n'en a eu aucune de favorable, il a dû donc attendre quelques semaines afin d'avoir sa première réponse favorable une situation angoissante qui s'est réélu, quelques jours après, avant le début des épreuves du Baccalauréat et s'est donc retrouvé dans une situation favorable et chanceuse mais combien d'étudiants subissent à la fois le stress des épreuves du Baccalauréat et le stress de sa mission Parcoursup Lisa 17 ans en 2022 avec d'excellents résultats au bac, elle souhaite faire une double licence en droit et en sciences politiques à Rennes, ville qui n'est pourtant pas dans son secteur, elle a donc été classée 2 millième sur la liste d'attente, l'accès à l'enseignement supérieur cristallise de nombreuses inquiétude et incompréhension au delà des questions immédiates sur la formation souhaité ou l'organisation de la vie étudiante se pose donc la question de l'avenir de nos jeunes, ils ont parfois le sentiment de faire des choix importants sans pour autant maîtriser tous les paramètres de leur décision pour tenter de répondre à ces enjeux, Parcoursup a été mis en place en 2018 en remplaçant en remplacement du dispositif Admission post-bac depuis son lancement, de nombreux élus, notamment au Sénat, on interpellé le gouvernement sur les difficultés rencontrées par les élèves et le et leurs professeurs lors de son utilisation sur l'opacité des algorithmes de la plateforme, ou encore sur l'anxiété provoquée par la procédure en ligne en septembre 2022 82 % des bacheliers déclaré avoir trouvé la procédure trop stressante, bref, après 4 années d'existence, le système demeure trop peu compréhensible et difficilement lisible, si l'on ne regrette pas les écueils d'admission post-bac, comme le tirage au sort, ou encore les files d'attente devant la fac ou le 1er arrivé était le premier inscrit le dispositif Parcoursup et plus largement l'orientation de nos élèves de terminale doit être repensé tout d'abord, je pense à l'accompagnement à l'orientation qu'il est la clé de voûte de la réforme du lycée, mais qui est le parent pauvre de l'Éducation nationale, avant même que les élèves ne n'inscrive ne s'inscrivent sur la plateforme, nous constatons un déficit de formation des professeurs, alors même que ce sont eux qui ont la charge d'accompagner leurs élèves dans leur orientation, selon la Cour des comptes en 2020 de nombreux professeurs et proviseurs déclaré n'avoir reçu aucune formation spécifique qui pourrait exercer leur missions d'orientation, les récents modules mis en place par les rectorats, à la suite de la loi d'orientation et la réussite des étudiants concerne principalement les points pratique et ceci au détriment de l'accompagnement et du conseil aux élèves dans leurs choix de formation et de métier, faire de l'orientation, une matière à part entière avec des accompagnants spécifiquement formés peut être une prise d'une piste de réflexion pour être plus efficace, ensuite les heures destinée à l'orientation intégré à la dotation horaire globale qui sert trop souvent dehors d'ajustement pour l'enseignement des spécialités, trop souvent, une fois les heures de spécialités d'options posées, il ne reste quasiment plus rien pour faire de l'orientation, ce système renforce les inégalités territoriales entre les établissements ayant une culture de l'orientation et d'autres moins mobilisé sur ces problématiques, il peut également être une source d'inégalité sociale avec l'émergence de coach privé en orientation, le passage du système d'admission post-bac à Parcoursup a fait passer les élèves d'une logique d'affectation et une logique de classement alors qu'Admission post-bac, demander à chaque lycéen un classement a priori de ses voeux pour l'enseignement supérieur Parcoursup met fin à ce système de hiérarchisation dès le début de la procédure, le lycéen doit désormais effectuer de nombreux choix sans pour autant indiquer ses préférences, son affectation semble davantage dépendre de sa place dans les classements de chaque formation que de son projet d'orientation ou de sa véritable motivation Parcoursup a conduit à la mise en place de plus de 15000 algorithmes remplaçant crises des critères objectifs nationaux et non académiques, en l'absence d'harmonisation nationale comment distinguer de dossiers scolaires construits par des enseignants dans des établissements différents et, selon des critères différents, les fortes disparités entre les différents lycées conduit certaines formations à prendre en compte les lycées d'origine des candidats pour effectuer leur classement sans que l'objectivité de la méthode ne soit garantie, nous sommes donc en droit de nous interroger sur la pertinence de certains critères d'évaluation, toujours selon le rapport de la Cour des comptes, il apparaît également que la bonne information des candidats sur les critères de classement des formations, quels ils prétendent n'est pas complète les attendus publiés ne semble pas toujours correspondent aux critères retenus par les commissions d'examen des voeux et souvent ces dernières utilisent des outils informatiques d'aide à la décision pour effectuer un pré-classement des étudiants, il convient donc de rendre publics les algorithmes utilisés afin que les dispositifs soient plus transparents, l'instauration de cette nouvelle procédure a conduit à un surcroît de travail très significative pour les équipes de l'éducation nationale, souvent pour des opérations administratives sans aucune plus Value pédagogique dans l'enseignement supérieur, ce sont des milliers d'enseignants qui examine des dossiers dans plus de 15000 formation enfin le dispositif Parcoursup n'a pas permis de réfléchir à des solutions pérennes face au défi que représente la massification de la population étudiante et à la nécessité d'accueillir ces nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions, en 50 ans, elle est passée de 20 % à 79 % sans autant de candidats potentiels voulant légitimement accéder à des études supérieures, alors qu'est annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif trouve ton master pour les étudiants peut postuler en master deux nous sommes inquiets, battu le suivre la même logique que Parcoursup 4 années après la mise en oeuvre de Parcoursup les bénéfices de la nouvelle procédure d'orientation sont difficiles à estimer aujourd'hui le taux d'échec à l'issue d'une première année d'études post-bac reste très élevé et concerne près d'un étudiant sur 2, particulièrement dans les filières non sélectives aussi nous nous félicitons de la mise en place d'une mission d'information sur le dispositif Parcoursup et nous suivrons attentivement ses travaux et ses conclusions, Madame la Ministre, l'éducation nationale ne devrait-elle pas aider les jeunes à trouver leur voie plutôt que les forcer à emprunter des voies sans issue, je vous remercie. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jean. Alors je ne peux pas répondre à tous, je vais d'ailleurs pas suivent ma fiche, j'ai vu lancer comme ceux-ci, mais d'abord je voudrais vous dire que nous avons tous des exemples d'Antoine Lucie je ne sais plus de cas particuliers ma difficulté à moi et ma mission, c'est de s'occuper de tous les étudiants, des cas particuliers uniquement, et c'est bien là une des difficultés, vous l'avez aussi dit alors effectivement l'accompagnement déserte des enseignants et quelque chose sur laquelle nous allons travailler cet accompagnement des enseignants qui veut dire, être à leur écoute, leur communiqué, les outils et des outils simples et faciles d'usage pour enseigner les et lycéens, nous y travaillons et vous le verrez dans mes propositions, je voudrais aussi rappeler la hiérarchisation des voeux cette hiérarchisation des feux qui n'est pas présente dans Parcoursup elle éviter sur APB l'autocensure d'APB, comme je le disais, un étudiant qui avait dit veut avant, hé bien, s'il était pris au 3ème 4ème veut ne savait même pas s'il pouvait être pris à ses autres veut ça veut dire qu'il décidé en février de d'un retour qu'il l'avait, en juin, juillet, août, septembre un jeune à 17 18 ans je pense pas que cela, enfin, c'est plutôt un progrès au niveau de Parcoursup, vous avez aussi parlé du stress induit, on le comprend ce ressenti de stress induit que nous avons amélioré et c'est là aussi un des facteurs d'amélioration que nous allons essayer de proposer dès cette année, avec mon collègue m'avez interpellé en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais en tant que ministre de l'enseignement supérieur, j'essaye de effectivement orienter les étudiants vers leur réussite et je peux vous dire que parcours pour le le la plateforme de master je je vous incite à les lire ce que je j'en disais parce que ça sera trop long à expliquer ici, mais elle n'est pas du tout basé sur les les principes de Parcoursup mais, comme dans Parcoursup, elle est d'abord passé sur un principe humain de commission d'examen des voeux des dossiers des étudiants par des enseignants dans le métier, la carrière et j'oserais dire toute leur vie et là pour la réussite de tous nos étudiants je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Bernard Phia l'air du groupe RDSE. J'ai monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'occasion de la dernière rentrée scolaire devant les recteurs d'académie, le président de la République a déclaré, je le cite nous rêvons d'une école qui fassent réussir nos enfants et qui fassent réussir la France oui, la réussite des enfants est à la fois une histoire individuelle et une amende collective qui mobilise d'importants moyens et des politiques publiques, qu'il nous faut sans cesse interrogé sans vouloir anticiper le très proche : examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2023, je soulignerai simplement qu'avec 59 7 milliards d'euros, l'éducation nationale consomme la part la plus importante du budget de l'État, si je mets de côté la mission remboursements et dégrèvements, un tel montant nous invite en effet à regarder de près ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce soir, il est question de débattre de l'orientation post-bac, une phase déterminante pour le futur de chacun de nos jeunes concitoyens dans l'imposant système de l'éducation nationale, quel bilan pouvons-nous tirer de Parcoursup après Craig 4 années de sa mise en oeuvre, si l'on s'en tient au chiffre publié sur la plateforme 836000 candidats concernés en 2022 3 millions huit de proposition d'admission et 93 % de lycéens contenté en face, principal à l'issue de la phase complémentaire, seuls 160 bachelier serait resté sans proposition, c'est peu, c'est mieux que l'année précédente, mais bien sûr, pour les familles concernées, c'est beaucoup, on observe toutefois que les commissions d'accès à l'enseignement supérieur jouent bien leur rôle dans l'accompagnement de ces élèves sans solution et j'en profite pour saluer leur travail. Parcoursup semble globalement fonctionné éviter certains écueils de l'ancien dispositif APB jugé à l'époque totalement déshumanisé et trop complexe, si les quotas d'affectation des élèves sont remplies, ce système d'orientation respecte-t-il un principe républicain fondamental, celui de l'égalité des chances dans l'accès aux études supérieures. Des orientations ne se ne serait-elle pas davantage subi plutôt que voulu 28 pour 100 des d'élèves se déclarent insatisfaits de leur sort d'admission dans le supérieur Parcoursup n'évite pas la sélection selon un rapport de la Cour des comptes de 2020 sur l'orientation des étudiants, certains de mes collègues l'ont rappelé la façon dont procèdent, la commission d'examen des voeux n'est pas totalement transparente la publication ex-Post des critères retenus à l'issue de la procédure d'inscription ne suffit pas à garantir un traitement de non-sélectivité. Si le Conseil constitutionnel a donné raison, secret des délibérations des jurys, il serait cependant souhaitable de définir certains des paramétrages retenus par la commission d'examen des voeux et d'en écarter certains je pense en particulier aux critères du lycée d'origine parfois utilisé pour le départage dans les filières non sélectives tension. Enfin, en amont de Parcoursup bien que l'article L 313 tirer un du code de l'éducation, affirme le droit au conseil en orientation, il est urgent de renforcer la phase d'information individualisée des élèves durant leurs 2 dernières années de lycée, les politiques publiques en la matière devrait notamment mieux prendre en compte les difficultés propres aux élèves des milieux socialement défavorisés, il existe un phénomène bien connu d'autocensure chez les élèves les moins favorisés quant à leur choix d'orientation par ailleurs plus de la moitié d'entre eux se retrouvent seuls à saisir leurs données sur Parcoursup contrairement aux élèves des milieux favorisés, dont les 2 tiers sont épaulés par leurs parents pour terminer mes chers collègues, je n'oublie pas le problème du stress, de plus en plus répandu chez les élèves, comme il vient d'être évoqué, il existait auparavant chez les lycéens, une sorte d'insouciance, dont on a

plutôt que la promesse d'une phase d'angoisse en effet tout comme APB Parcoursup suscite encore beaucoup d'inquiétudes et chez les parents aussi mercredi dernier le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a rappelé devant la commission Culture éducation l'importance du bien-être à l'école et je partage sa préoccupation, Madame la Ministre, vous le savez depuis la pandémie, l'attente est immense sur cet aspect de la vie scolaire qui n'est pas suffisamment pris en compte par conséquent mon groupe RDSE compte sur vous pour la mise en oeuvre de politiques visant à redonner aux jeunes l'espoir de tous les possibles. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Si monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bernard à l'air, croyez-le bien, pardon je partage comme vous. Cette ardente obligation de faire réussir nos étudiants, de l'égalité des chances et de l'accès à l'enseignement supérieur et aussi pour tout cela, l'obligation de la transparence, non comme un outil pour pour forcer des enseignants qui profiteraient dit-on de l'opacité pour faire une sélection discriminante mais parce que je crois comme vous que la transparence peut être un levier pour améliorer l'accompagnement à l'orientation pour rendre les résultats de Parcoursup plus plus prévisible et au final pour réduire ce stress ressenti du stress des lycéens et nous allons-y travailler en ce sens Parcoursup a accompagné depuis 5 ans, les formations pour aller vers plus de progrès dans la compréhension de ces critères d'analyse des candidatures, là où il n'y avait rien, nous avons créé des attendue, puis l'obligation d'afficher les critères et nous irons plus loin comme je l'indiquerai tout à l'heure dans ma réponse finale approfondir la transparence évidemment oui, mais comme vous l'avez dit, je tiens aussi à préserver ce secret des lits délibération collégiale des enseignants, ce n'est pas un réflexe corporatiste et encore moins la volonté de sauvegarder l'opacité, mais c'est la conviction que la délibération des enseignants est un acquis, comme vous l'avez rappelé que le Conseil constitutionnel a reconnu et la garantie d'un regard humain l'auto mais l'automatisation que la CNIL avait d'ailleurs reprochait à APB, ne tombons pas collectivement dans cette caricature qui jettent l'opprobre sur injustement sur les milliers d'enseignants qui font l'examen des dossiers avec détermination et la volonté chevillée au corps d'accueillir et de faire réussir leurs futurs étudiants, je voudrais rappeler la volonté de la loi hors de Parcoursup pour les étudiants boursiers les favoriser la prise en compte des cordées de la réussite et tout l'accompagnement que je vous présenterai sur les enseignants du secondaire et aussi les parents d'élèves, il y aura aussi un axe de travail : je vous remercie et il y aura des progrès à faire et qui seront fait merci. Merci madame la ministre et la parole est maintenant à notre collègue Max Brisson et le groupe, les républicains. Ce président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais remercier le groupe CRCE pour ce débat, et salué l'intervention gaullienne de Pierre Ouzoulias tout à l'heure en 2000 19 au Sénat mais Jean-Michel Blanquer, a déclaré à propos de Parcoursup et de la réforme du Baccalauréat pour la première fois un véritable pont s'est construit entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire, 3 ans après ce pont est-il véritablement en place, on peut en douter, pourtant en 2018, 2019 une opportunité sans précédent se dessiner le mécanisme APP était à bout de souffle et Parcoursup paraissaient s'imposer pour apaiser l'entrée dans le cycle des études supérieures, avec le système d'orientation ou le dossier de l'élève et donc ses capacités étaient davantage considéré au fond Parcoursup apparaissait comme le moyen de renouer avec une école méritocratique à un moment où beaucoup de parents crier leur inquiétude de voir leurs enfants dans l'incapacité de prendre un ascenseur qui ne les avait pas eux-mêmes conduit là où notre société leur avait au moment laisser espérer une place, c'est bien dans ce contexte qui est intervenu, la réforme de Parcoursup puis celle du Baccalauréat et là, c'est bien dans ses torts de que la réforme a été conduite malgré les nombreuses alertes qui étaient alors lancées sur l'inversion du calendrier des réformes à l'origine d'effort majeur devaient porter sur l'orientation, 3 ans après, le constat est implacable, comme l'ont montré tout à tour Sylvie Robert et Jean ANG la dotation horaire qui lui est consacré est insuffisante, bien souvent, ces heures sont utilisés pour terminer les programmes de plus et professeurs, manque de formation et parfois d'pour accompagner les élèves dans leur choix de spécialité et leur poursuite d'études, si la réforme est inachevé, c'est pas ce qu'au lycée, elle ne s'est pas donné les moyens de sa réussite de même elle c'est très inégalement pencher dans la du Mans supérieur qui peinent à s'adapter, on constate qu'en dehors de quelques associations de spécialités qui débouche sur des parcours construit de poursuit des études, les spécialités du lycée restent mal articulé avec les formations de l'enseignement supérieur, peu de partis minoritaires des établissements d'enseignement supérieur ont en effet réellement anticiper la réforme pour prendre en compte des profils plus diversifiée à l'opposé, la plupart à temps pour agir, l'arrivée de la première cohorte de lycéens ayant éprouvé cette réforme sur la totalité de leur scolarité dans le secondaire, plus grave encore dans de nombreux formation supérieure les résultats du tronc commun sont davantage mis en avant que les spécialités cela va l'encontre de la réforme, cela lui tourne le dos en effet l'un des objectifs était de faire émerger des parcours plus personnalisés, incarnée par le choix de spécialité avec un objectif essentiel, celui de la plus grande réussite des étudiants dans le supérieur, le fossé entre le sud et le Scot est définitivement consommée lorsque l'on sait que plus de la moitié des élèves abandonnent entre la première et la terminale des spécialités comme sciences de l'ingénieur ou numérique et sciences numériques par crainte de ne pas être pris en classe préparatoire, alors même que les écoles d'ingénieurs sont désireuses de ses spécialités, c'est là que l'on mesure l'échec de la réforme, elle ne me permet pas aux lycéens, ce qui était pourtant son but original de se muer progressivement d'étudiants et de se donner un maximum de chances, c'est là que l'on mesure l'échec du continuum lycée licence, c'est là que l'on constate que le pont qui évoquait Jean-Michel bancaire entre l'enseignement secondaire et le supérieur est loin d'être achevée, et c'est donc à l'aune de cet échec qu'il faut analyser les angoisses des futurs étudiants adore famille face à Parcoursup les débats autour des algorithmes mais du fonctionnement technique de la plateforme, les émotions autour des lycéens sans solution ou du manque d'accompagnement sont d'abord le résultat des faiblesses de l'articulation entre la réforme du Baccalauréat et les attendus de l'enseignement supérieur, certes des progrès doivent être faits sur le fonctionnement de la plateforme, mais l'essentiel réside dans une approche plus large et plus volontariste de l'orientation des lycéens, une réelle prise en considération du nouveau Baccalauréat par l'enseignement supérieur dans la définition de ses attendus et en effet, au delà des enjeux inhérents à la plateforme Parcoursup et à son fonctionnement, c'est bien le continuum lycée licence bac moins 3 bac plus trois qui reste à construire, c'est le pont dont parlait Jean Michel bancaire qui reste à constituer, alors Madame le Ministre, comment envisagez-vous au delà des amélioration du fonctionnement de la plateforme à travailler avec votre collègue de l'Éducation nationale à construire ce continuum et un système d'orientation qui permettent de manière apaisée, a des il de trouver dans l'enseignement supérieur, l'approfondissement de leur choix fait au lycée. Merci, cher collègue, la parole à Madame la Ministre. Si, pardon, merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, les sénatrices. Alors tout d'abord, vous avez évoqué, avec raison, l'enjeu de la continuité des parcours entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur je voudrais d'abord vous dire que c'est une question qui m'anime depuis des années aussi, au fond, je vous dirais que c'est l'un des grands défis de notre temps de temps d'avant et de temps, d'aujourd'hui et de demain, car ce qui se joue, c'est bien effectivement une meilleure orientation dans le secondaire, pour sécuriser les parcours des lycéens, mais aussi, et vous l'avez dit, une plus grande personnalisation des parcours dans l'enseignement supérieur pour favoriser la réussite des étudiants pendant longtemps le moins trois, plus trois est resté un concept, une coquille vide ou quelque chose que l'on essayé d'atteindre avec Parcoursup la réforme du lycée, nous avons ouvert la voie à cette continuité, moins trois, plus 3 pour éviter ces ruptures et je peux vous dire qu'avec Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, nous avons décidé d'y travailler et de franchir un pas et là je pose mes fiches je voudrais vous répondre parce que je pense que ce que vous me dites, et je vais voir le résumé, c'est une philosophie de l'enseignement que nous devrions discuter, c'est que nous sommes au XXIe siècle, vous avez parlé du numérique, vous avez parlé du digital, je pourrais faire pour vous parler des sciences pour l'ingénieur de. Beaucoup, beaucoup de discipline ou de compétences ou de connaissances dont ont besoin nos jeunes aujourd'hui et je pense que c'est plus qu'aujourd'hui que de revoir la continuité du moins trois, plus trois, même si elle est nécessaire et nous devons y travailler, c'est une philosophie de comme dirait Montaigne de savoir si il faudrait une tête bien faite ou bien apprendre à apprendre et je peux vous dire oui, je peux repenser de ce dont a besoin, nos élèves et nos étudiants tout au long de leur parcours tout au long de leur métier en connaissance et en compétence que nous devons apprendre au lycée à à l'université, dans les écoles, je pense que c'est un travail de fond que nous devons mener dans le cadre du moins trois, plus 3 mais dans le cadre d'un enseignement pédagogique du XXIe siècle avec des passerelles et avec une formation qui doit être une formation tout tout tournant de la vie et c'est une refonte complète que nous devons repenser, non seulement dans le moins trois, plus trois, je vous remercie. Merci madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Pierre de colle pour le groupe, les indépendants.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en les mineurs à pour l'intervention je veux remercier le groupe CRCE pour ce débat, depuis sa création en mars 2018, la plateforme Parcoursup contribue à une refonte bienvenue du système éducatif français, il vise à répondre aux difficultés d'accès aux études supérieures, après 4 ans d'exploitation la plateforme continue à répondre à la mission que le Parlement et le gouvernement lui ont confié, mais des ajustements reste nécessaire, quant au délais de réponse et la lenteur des processus d'affectation, pourtant, la prise en compte des inégalités subies par les jeunes au bureau reste le parent pauvre de de nos politiques publiques, selon les données du ministère de l'Éducation nationale 10 millions de jeunes de moins de 20 ans grandissent dans des communes de moins de 25000 habitants, comme l'a montré le sociologue Nicolas relaye l'enclavement à ses conséquences réelles sur les opportunités offertes aux jeunes, bien souvent, ils doivent se restreindre formation proposées sur les territoires, ou bien partir d'autres raisons parfois difficilement quantifiable, explique les difficultés d'accès aux formations post-bac, c'est notamment le cas de l'autocensure, le manque d'information disponible il y a des difficultés économiques, ainsi que l'ensemble des freins à la mobilité divers en octobre 2018, le gouvernement avait lancé une mission visant à mieux prendre en compte les particularités de certains territoires, en particulier les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux, c'était une bonne chose, plusieurs conclusions s'imposent d'une part les politiques scolaires rural ont tendance à être parcellaire et mal articulé avec les politiques d'aménagement, d'autre part, les inégalités territoriales se creusent si le zonage de scolaire prend seulement en compte les difficultés sociales concentrera même territoire, il oublie de ce fait, les difficultés disperser la mobilité ou la fracture numérique, par exemple, trop souvent les inégalités scolaires ne sont appréhendés que sous l'angle des inégalités sociales, mais n'oublions pas les inégalités territoriales sujets auquel nous sommes attachés dans cette maison, mes chers collègues, c'est notamment le cas avec la rubrique centres d'intérêt, complété par les jeunes futurs étudiants pour augmenter leurs chances d'intégrer la filière de leur choix, cette rubrique est source d'inégalités face à la demande croissante et au caractère non extensible des locaux universitaires, certaines écoles sont en effet tentés de sélectionner les étudiants sur des critères dépassant le simple dossier scolaire dès lors deviennent parfois nécessaire des séjours linguistiques à l'étranger, un service civique ou encore le BAFA, autant de facteurs censés permettre aux jeunes de se démarquer des autres, or les jeunes des territoires ruraux ne dispose pas des mêmes ressources que ceux des grandes agglomérations, ils sont trop souvent démunis lorsque vient le moment de compléter leur profil sur la plateforme, l'accueil a et l'accès par un stage à une activité extra-scolaire ou encore à une association dans laquelle s'engager et bien évidemment plus facile en zone peu denses, là encore, les origines géographiques restent déterminantes dans l'orientation post- bac et dans la difficulté et la capacité à se projeter dans l'avenir, en octobre 2022 l'enquête une jeunesse engagée sur les étudiants de Sciences Po a été publié pour 36 % d'entre eux, ce sont les relations qui compte le plus dans la formation de l'élite, contre 20 % en 2002 les diplômes sont déterminants pour seulement 14 % d'entre eux, contre 36 % en 2002, cette étude doit nous alerter l'avenir est quelque chose qui se surmonte on ne le subit pas, on le fait, disait Georges Bernanos à l'auteur que j'affectionne tant il s'est attaché à décrire les charmes de ma région, les Hauts-de-France nous devons dessiner une politique éducative, prenant en compte l'ensemble des jeunes leur parcours et leur territoire d'implantation, il faut pour cela compléter des dispositifs actuels d'égalité des chances parcoursup dont l'algorithme détermine le parcours de notre jeunesse doit pouvoir y contribuer, les jeunes ruraux demande tout simplement à bénéficier des mêmes chances de réussir que les autres, à nous de montrer à notre jeunesse rurales comme urbaines que nous avons entendu cette demande et que nous la prenons à bras le corps, il est crucial en effet que chaque jeune Français, d'où qu'il Vienne bénéficient des mêmes chances lors de son orientation post-bac, dès lors, Madame la Ministre, j'émets le souhait au nom du groupe, les indépendants que la fracture territoriale soit davantage prise en compte par la plateforme Parcoursup afin qu'elles contribuent à la réduire, je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre.

D'abord, merci, merci d'évoquer ce soir avec l'engagement que nous vous connaissons cette question de la fracture sociale et de l'égalité d'accès aux services publics pour les jeunes et en particulier, vous l'avez dit, pour les jeunes des territoires ruraux, une petite précision que vous m'accorderez non ce n'est pas un algorithme Parcoursup qui fait ou défait l'avenir de la jeunesse près, je l'ai dit précédemment, c'est bien le côté humain qui est présent dans cette procédure mais je vous rejoins complètement Parcoursup, comme les autres dispositifs qui est portée par mon ministère et celui de l'éducation nationale doit être mobilisés pour assurer l'égalité d'accès et de réussite pour tous les jeunes parcoursup y contribue, croyez-le bien, d'abord en permettant à tous, quel que soit le lieu d'habitation, d'accéder à la même information sur toutes les formations de l'Hexagone, je vous rappelle aussi que nous donnons avec Parcoursup une visibilité sur le réseau des BTS ou encore des IFSI dont on sait que leur maillage enfin permet de répondre aux problématiques d'attractivité des territoires ruraux pour lutter contre cette autocensure nous avons promu les cordées de la réussite en demandant précisément à ce qu'elle puisse concerner aussi les territoires ruraux, aujourd'hui c'est 26000 jeunes collégiens en collèges ruraux qui participent à ces cordées et seront sans doute mieux demain préparer au choix sur Parcoursup avec un accès favorisé, nous prendrons mieux en compte cet accès des cordées et des boursiers, mais pour répondre à votre problématique, vous le savez bien, il faut dépasser effectivement le seul cas de Parcoursup car les inégalités territoriales ne sont pas créés uniquement par Parcoursup c'est pour cela que ma prédécesseuse a mis en place avec le soutien des collectivités territoriales, ces Campus connectés qui permettent d'associer études à distance et soutien à la réussite de proximité, il y en a aujourd'hui 80 sur le territoire et nous allons continuer à travailler sur le maillage du territoire avec des formations présentiel tellement nécessaire à nos étudiants, je vous remercie. Merci madame la ministre et la parole est maintenant à notre collègue Jacques Grosperrin pour le groupe, les républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je remercie le groupe CRCE et Pierre Ouzoulias d'avoir mis en place, débat en tout cas de Parcoursup qui n'est-il pas celui de la question de la sélection, l'université, ses modalités, ses acceptabilité ses stigmates, en tout cas la hantise pour un gouvernement d'une loi Devaquet bis en 86 qui est encore dans toutes les mémoires des élus et de nous même un 1000000 dans la rue, sur 50000 pour la police et pourtant les défis restent les mêmes, je disais, je disais, déjà en 2018 lors du débat sur la loi alors que les étudiants étaient de plus en plus nombreux avec un échec massif en licence et c'est ainsi que les difficultés d'APB en 2017 ont précipité les choses et imposer qu'une réforme de l'admission de l'enseignement supérieur soit menée dans l'urgence suite à un tirage au sort inacceptable, fallait-il pour autant comme je disais, j'ai été appelé avec l'eau du bain car bien trop disait déjà à partir de 2008, un portail de coordination des admissions dans l'enseignement supérieur, ce qui faisait dire à l'époque à la Cour des comptes qu'il fallait une véritable simplification pour gérer les flux, sans être un système d'orientation ou ni un instrument de sélection, ce n'était pas pour la Cour des comptes, le signe d'une défaillance intrinsèque de l'outil, mais un révélateur des choix ministériels en matière d'accès à l'enseignement supérieur qui ne répondait pas à la réalité de la situation est-ce que cela changer Madame la Ministre, ce sera ma première question un travailler avec les universités, les branches prol et les conseils régionaux doit être menée avec les rectorats afin de réorienter l'offre de formation, il faut aussi l'adapter aux besoins présents et futurs de notre économie, la CMP, du 13 février 2018 au Sénat où Gabriel Attal rapporteur pour l'Assemblée nationale et moi-même pour le Sénat comme rapporteur et vous tous collègues présents qui avait déjà formulé de nombreuses inquiétudes reste d'actualité et je la mesure mais notre sens des responsabilités pour une CMP conclusive allait peser car 850000 jeunes étaient en attente de Parcoursup avec une loi promulguée promulgué le 8 mars 2018 pour une rentrée, 6 mois plus tard, et certains sur ces bancs se souviennent il a pas simplement les élus sénateurs aujourd'hui les problèmes restent les mêmes, car la massification de la formation post-bac et la démocratisation soulève de difficultés, le fonctionnement, il s'agit tout simplement des capacités d'accueil des moyens avec une dépense pour l'enseignement supérieur qui atteint juste 1 virgule 5 % de sa richesse, la France est très loin des 2 % du PIB fixé par le Livre blanc et le 2ème point c'est l'équité et l'efficacité d'un système l'inégalité d'accès et de réussite qui est aujourd'hui largement renseigné alors que le diplôme reste la clé d'accès à l'emploi que sa valeur performative augmente avec le niveau d'étude et que les grandes écoles restent gagnante dans ce contexte général Parcoursup reste le symbole de nos objectifs, aussi bien que de nos limites et parfois insuffisantes, mais il a permis néanmoins un meilleur effort collectif d'orientation et une information plus lisibles, cela favorise, a une responsabilité accrue des étudiants sur ce qui sera attendu de les critiques ont été trop nombreuses, et puis l'origine système trop concurrentiel lenteur efficacité insuffisante, absence de transparence et pourtant le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité du dispositif d'accès à Parcoursup le 3 avril 2020, chaque établissement d'enseignement supérieur doit être en capacité de rencontre des critères en fonction desquels sont examiner les candidatures dans le cadre de Parcoursup à stabiliser juridiquement Parcoursup et légitimer le travail des universités sur ces bases de stabilisation, il est difficile d'imaginer la suppression de la plateforme, même si plusieurs candidats lors des présidentielles, avait proposé la suppression, mais quelle solution alternative sur ce débat sur ces bases, plusieurs questions émergent, où en est-on aujourd'hui quelles pistes pour mieux gérer 2023 quel objectif chiffré pour la prochaine rentrée prochaine phase de The quels indicateurs fiables sur l'efficacité du système quelles pistes d'évolution sur liste d'attente et des lycéens qui se retrouvent sans affectation, comment assurer enfin une place pour tout autant de questions qui génère chez nos une vision négative ou déformée de Parcoursup avec un baromètre de confiance qui montre une réelle désillusion qui ne permettrait pas un accès équitable aux supérieur 36 % reste très indécis insatisfaits des délais réponse des propositions d'admission le fonctionnement même de la plateforme qui impose un travail en amont difficile pour beaucoup, le processus de validation qui peut conduire à une forme d'autocensure, poussé à l'extrême, enfin comment remédier à cet axe critique qu'elle peut être vos propositions, Madame la Ministre, les inégalités réelles si lutter contre les inégalités ressenti communiqué me davantage Parcoursup prend-il suffisamment en compte ses complémentarités, c'est aussi toute la question de la mobilité des jeunes un nombre accru de lycéens quittent leur région pour étudier des quotas ont été mis en place, imposer, bien sûr, notamment pour les établissements de la capitale, bilan Chive perspective et conséquences de cette mobilité, ce sera le rôle et la fonction de notre mission, la responsabilité de notre cher Max Brisson qui sera effectué au Sénat avec l'ensemble de tous les sénateurs, ici présent, je vous remercie.

un petit peu en vrac à vos réponses, mais quand même, quel progrès apportés par Parcoursup je vais le redire aujourd'hui, il y a plus d'admission les les évolutions et les améliorations continues sont réels, même si, et je le redis, il doit y en avoir encore pour moins de stress, plus d'accompagnement plus d'accès mais 93 % des lycéens ont au moins une proposition aujourd'hui, c'est le chiffre qui les montre, et c'est une réalité. Des candidats ont sont accompagnés tout au long de procédure, je voudrais rappeler qu'il y a 11 campagne téléphonique qui appelle en SMS ou au téléphone, les candidats un par un à à partir d'un moment donné au niveau de Parcoursup le travail des cas est-ce qu'on a salué, que je salue et à la fin, effectivement 160 lycéens étaient encore à la fin de la procédure, mais continue à être accompagné en fin de procédure, il en restait, il n'y a pas longtemps 33 sans proposition d'accès nous n'arrêtons pas après les caisses et puis les rapports publics je rappelle aussi pour avoir des chiffres pour avoir ces critères de transparence en 2022 ça sera 11732 rapport public que l'on a reçu aujourd'hui et que qui seront rendus publics sur Parcoursup et qui seront utilisées dans la suite pour les étudiants pour les orientations donc de même pour la lutte contre les inégalités, 5 points de plus pour les boursiers, on l'a vu, de 20 à 25 pour 100 de boursiers et beaucoup plus de mobilité avec un accompagnement de 500 euros pour les boursiers pour avoir de la mobilité et je le redis, l'idée de l'accès, c'est l'idée de l'accès en 1er cycle en proximité mais aussi l'idée d'accès, de ne pas interdire à un étudiant d'accéder partout en France, à à la formation qu'ils souhaitent et dont il peut avoir accès, je voudrais vous redire un point avant de terminer vous parlez beaucoup, tous, de l'échec massif en licence, c'est une réalité, on le sait, mais on est bon, on est mauvais, c'est toujours par rapport à quelque chose et je voudrais vous inciter à regarder le dernier rapport de l'OCDE qui nous permet de nous comparer par rapport aux formations à l'Europe, ah ces échec en 1er cycle à ce 2 % de PIB et comment la France et son enseignement supérieur par rapport au PIB des pays permet de se positionner aujourd'hui oui, il y a des progrès à faire, mais vous verrez que, quand même, même par rapport aux établissements européens, nous tenons notre place merci beaucoup. Merci madame la ministre, et pour terminer ses interventions, la parole à notre collègue Stéphane Piednoir du groupe, les républicains. C'est le président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour mettre en perspective nos débats du jour et pour conclure, permettrait de, de faire un peu d'historique, comme chacun sait, le Baccalauréat est à la fois le 1er, diplôme de l'enseignement supérieur, mais également le sésame pour accéder à ce niveau, chaque année, ainsi plus de 600000 jeunes bacheliers aspirent à une poursuite de d'étude qui correspondent à leurs ambitions et si possible à leur capacité, tout le monde peut comprendre que cette grosse machine nécessite un minimum d'organisation pour être efficace pour relativiser les griefs qui peuvent être légitimes sur le système actuel, je voudrais évoquer un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître beaucoup d'entre nous ont connu une procédure d'affectation avant l'heure du du numérique qui consistait pour les filières dites sélectives a envoyé son dossier par la Poste à l'établissement accueillant la formation de son voeu préférentiel puis en cas de réponse négative, toujours par courrier répéter la procédure pour chacun, des voeux suivant rigoureusement cher cher Pierre, cela s'appelle un algorithme, et vous conviendrez qu'il n'était pas optimale, y compris sur le fond puisque aucune justification du refus n'était exigible depuis la massification de l'accès au Baccalauréat, la croissance quasi-ininterrompue du taux de réussite et la multiplication des cursus Post bac ont considérablement alourdi la tâche de ceux qui sont chargés d'examiner les dossiers et de faire en toute conscience professionnelle, les choix d'affectation, un système entièrement Manuel n'était plus tenable et nous avons vu l'apparition de l'admission post- bac qui assure répondent globalement, quoi qu'on en dise, à cette situation. la difficulté porte sur le problème théorique, dit des mariages stable consistant à trouver étant donné, N O mais femmes et leur liste de préférence une façon stable, de les mettre en couple, c'est l'algorithme de gueule et chapelets qui, en 62 parvient à résoudre ce problème qui servira pour élaborer la plateforme Admission post-bac, mais il y a un biais majeur, la fonction de préférence qui privilégie un groupe plutôt que l'autre, le parti pris pour admission post-bac, comme pour Parcoursup d'ailleurs, qui reprend les mêmes caractéristiques techniques, c'est de donner priorité aux préférences de l'établissement. Qu'est-ce qui nécessitait une refonte de cette procédure essentiellement la hiérarchisation des voeux et leur grand nombre, compte tenu de la multiplicité des combinaisons possibles les grandes nouveautés de Parcoursup institut avec la loi, orientation et réussite des étudiants en 2018 sont l'extension de la procédure aux universités et à plus de 15000 formation ainsi que la publication d'attendu pour mieux informer chaque candidat et le diriger vers les choix les plus pertinents, mais beaucoup reste encore à faire en termes d'orientation et c'est sur ce point que j'aimerais insister. Comme l'avait pointé la Cour des comptes en 2020, l'orientation des élèves est identifié comme une priorité des pouvoirs publics, mais la mise en oeuvre de cette politique rencontre des obstacles majeurs la stratégie d'orientation dans le supérieur, commence sans doute plus tôt aujourd'hui qu'il y a plusieurs années et le fait même d'évoquer une stratégie laisse entrevoir toutes les difficultés auxquelles peuvent être confrontées certains jeunes et leurs familles, les inégalités sociales se creusent donc au niveau bac moins trois puisque les milieux les moins favorisés se repose quasi intégralement sur les équipes éducatives pour rendre pour prendre en charge l'orientation de leurs enfants, pour répondre à cela, la Cour des comptes et l'inspection générale de l'Éducation pointe un besoin croissant en matière d'information et de professionnalisation des différents acteurs du processus d'orientation, cela vaut pour les établissements scolaires mais également pour les formations de l'enseignement supérieur dans leur processus de recrutement, nous espérons, Madame la Ministre, que des actions des actions concrètes seront entreprises dans ce domaine pour permettre à Parcoursup d'atteindre l'un de ses objectifs essentiels mise en avant en 2018, Merci, la parole à Madame la Ministre, vous pouvez répondre à monsieur Piednoir mais on vous pouvez si vous le souhaitez, enchaîner sur la réponse globale puisque, ensuite, de toute façon je vous repasserai la parole pour faire la conclusion globale du débat, donc vous pouvez enchaîner les deux si vous le souhaitez. Merci monsieur le président je pense que je vais accepter parce que mes réponses dans la. Bilan global répondra probablement enfin certainement ah monsieur le sénateur noirs, donc si vous si vous le permettez, je peux vous répondre en même temps sur l'ensemble des réponses, ce qui permettra d'avoir une vision plus globale. Allez-y à allez-y.

prendre. Merci monsieur le président, et mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs. Alors permettez-moi tout d'abord vraiment de vous remercier de remercier pour ce débat pour la qualité de vos interventions, ce soir et tous les points pertinents, bien évidemment, et identifié que vous avez soulevés, je l'ai dit. Parcoursup n'est qu'une plateforme mais une plateforme qui doit être au service des futurs étudiants sur cette plateforme, les formations ont une responsabilité première, bien évidemment, au fond, ce qu'il faut rappeler au moment de clore ce débat, c'est que la procédure Parcoursup assure un échange entre les lycéens et entre les enseignants des formations post-bac avec l'aide, et c'est fondamental des professeurs principaux qui sont au plus près des lycéens, la loi du 8 mars 2018 la organisé autour de plusieurs ambitions qui sont, et je n'en doute pas partagé sur tous les bancs de cet hémicycle, l'ambition de renforcer l'accompagnement à l'orientation au lycée pour en faire un tremplin vers cet enseignement du supérieur, l'ambition de mettre fin aux inscriptions, par ordre d'arrivée, comme vous l'avez dit, dans la nuit ou par tirage au sort en fixant des règles transparentes, j'y reviendrai connue de tous, l'ambition aussi d'améliorer la réussite de tous les étudiants. L'ambition, enfin de renforcer la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur sur chacun de ces points, que de chemin parcouru quand même depuis 5 ans au lycée, l'accès à l'enseignement supérieur est devenue un enjeu majeur qui mobilise toutes les équipes éducatives, avec le souci de sécuriser, mais aussi d'accompagner le parcours des lycéens en 2022 plus de bacheliers ont eu de proposition d'admission et ils les ont eu beaucoup plus vite, comme le montrent les enquêtes et les différents chiffres et du supérieur, le nombre de lycéens sans solution à la fin de la procédure a été considérablement réduit au cours des années, ils étaient comme je l'ai déjà dit 100 60 en septembre 2022, et nous avons continué à les encadrer à les suivre pour réduire encore parce que chaque étudiant est important pour tous en 2023 en intégrant dans le dossier Parcoursup les notes des épreuves finales des enseignements de spécialité nous redonnerons toute sa légitimité au Baccalauréat, nous renforcerons l'objectivité de l'analyse des candidatures, mais aussi l'articulation, moins trois, que Parcoursup a fait progresser comme jamais auparavant la transparence, vous l'avez tous se rappeler est un objectif majeur au service de l'orientation des lycéens, nous avons encore des progrès à faire mais jamais autant de données n'ont été rendus publiques par mon ministère, les règles de Parcoursup sont simples et public : l'obligation faite aux formations de rendre compte de leurs critères et de leur choix est effectif pour cette session 2022, 11732 rapports ont été remplis par les chefs d'établissement et nous les rendrons tous accessibles, le tirage au sort, c'est terminé depuis 5 ans et l'automaticité que la CNIL avait reprochait à APB est fini, cessons d'affirmer qu'avec Parcoursup, la sélection se serait accru à l'université, oui, les règles d'admission ont évolué oui l'examen des dossiers et la règle parce que cela sert la méritocratie, mais aussi la réussite de nos étudiants in fine cette réussite étudiante, elle a progressé depuis Parcoursup d'au moins 5 virgule et cela sans tenir compte des résultats sans doute exceptionnel de l'année 2020, la tendance est claire et la personnalisation des parcours doit devenir et devient une réalité dans les universités, la démocratisation, enfin, a également progressé de 2000 depuis 2018, comme l'a plusieurs fois souligné le comité éthique et scientifique de Parcoursup, c'est plus 5,2 lycéens boursiers admis, c'est plus de mobilité étudiante c'est un accès renforcé des bacheliers professionnels et technologiques dans les filières professionnalisantes et bien sûr cette dynamique d'amélioration doit se poursuivre, c'est mon engagement : celui du président de la République qui a pris l'engagement, je cite, je cite, de Parcoursup, plus prévisible en donnant des résultats précis des années précédentes et en accompagnant mieux les familles avec le ministre de l'Éducation nationale, nous souhaitons prendre en compte le ressenti des lycéens et malgré une appréciation positive globale sur l'expérience parce que Parcoursup ils manifestent effectivement encore des attentes en terme de réduction du stress de transparence de la procédure, c'est pourquoi nous conduiront des améliorations qui s'articuleront autour de 4 axes stratégiques qui seront alimentés par plusieurs éléments de notre discussion de ce soir tout d'abord renforcer l'accompagnement à l'orientation pour aider les lycéens et leurs familles à faire des choix et favoriser la réussite des étudiants ensuite rendent l'examen des candidatures plus transparent et les résultats d'admission sur Parcoursup plus prévisible en 3ème axe : améliorer l'efficacité de la phase principale pour réduire l'attente des candidats et le stress induit il y a Max enfin prolonger le continuum de réussite du lycée vers l'enseignement supérieur pour favoriser cette réussite étudiante mais aussi l'insertion professionnelle après le cycle licence ces progrès nous les engagerons en lien avec les acteurs de l'enseignement supérieur, car rien ne pourra se faire sans celles et ceux qui donnent de leur temps pour les journées portes ouvertes pour l'examen des candidatures sur Parcoursup, et dont je sais pour avoir été l'une d'entre eux, qu'ils n'ont qu'un seul but : accueillir les futurs étudiants les former et les faire réussir dans leurs études et tout au long de leurs études, c'est normal que dans une période de choix, nous devons tout faire pour que ces choix se fasse dans la sérénité et ces processus sont en train d'être étudiée avec le ministre-dans l'enseignement supérieur pour être mise en oeuvre dès cette année et j'espère pouvoir venir vous les présenter dans le détail et l'année prochaine, lors d'un bilan vrai une vraie amélioration de ce système Parcoursup dans les chiffres disent déjà beaucoup et dans le bilan l'année prochaine sera encore meilleur, je vous remercie. merci, madame la ministre, et pour conclure le débat, je vais passer la parole à Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen avant de vous passer la parole, chers collègues, je voudrais rappeler à tous mes hein tous les collègues qui ont participé à ce débat que compte la ministre utilise son droit de réponse à chaque intervenant vous avez la possibilité d'une réplique d'une minute, personne ne l'a utilisé ce soir mais c'est parce que nous tous les ministres ne répondent pas systématiquement la question donc on a du mal à ce que les règles voilà à s'approprier toutes les règles, mais je le rappelle, parce que ça peut servir pour d'autres débats compte la ministre répond : vous pouvez aussi utiliser une réplique d'une minute à la suite de sa réponse pour conclure le débat Pierre Ouzoulias. Merci monsieur le président, la Ministre mais mes chers collègues, je voudrais très sincèrement vous remercier par pour la qualité de

pour vos réponses toujours extrêmement argumenté, et vous avez parfaitement illustré, ce qui est la la la dispute universitaire un échange rationnel sur sur des bases qui sont connaît tout le monde France université qui nous ont envoyé des notes extrêmement utile qu'on qu'on nourrit aussi nos nos nos discussions le point important pour commencer sur les consensus et je vais essayer de de présenter la plus honnête possible un certain nombre des des points des points sur lesquels nous sommes d'accord, chers collègues, le 1er point c'est vous avez rappelé ici avec force, mais c'est pas la première fois, votre souci d'illustrer une université républicaine c'est un c'est quelque chose de de tout à fait fondamental et nous pensons qu'à l'échelle internationale, le modèle français de l'école républicaine de l'université républicaine est un modèle d'avenir en dehors d'autres modèles de du modèle anglo-saxon par exemple qui est fondée sur d'autres, d'autres principes j'ajouterais puisque il a été question à plusieurs reprises d'égalité des chances que le service public repose sur l'égalité des droits, ce qui est pas tout à fait la même chose et ça une valeur, beaucoup, beaucoup plus important dans dans tous les deux bah finalement il y a plusieurs questions extrêmement importantes qui sont, qui sont revenus et qui, et qui n'ont jamais été réellement posées notre société, c'est-à-dire combien la France veut-elle d'étudiants aujourd'hui et qu'est-ce que la nation est prête aujourd'hui à à financer pour son université, question de fond qu'est ce que nous voulons, et je pense que ça, ça serait nettement plus intéressant de commencer par par ce débat là, on le voit bien, ces jours derniers que la question des mathématiques, a été tout à fait essentiel et hier, je crois, le PDG du CNRS a lancé un cri d'alarme en disant qu'il manquait de mathématiciens pour que la France pour que le CNRS continue à être à son niveau, là je pense qu'il nous faut nous poser ces questions pas filière par filière, mais par grandes masses de discipline est ce qu'on a encore besoin d'archéologue, ce qu'on a encore besoin d'historiens, c'est ce je, je, je crois que c'est tout à fait important de placer le le débat à ce niveau-là, parce qu'ensuite on peut réfléchir sur les modes de recrutement, les procédures de recrutement, mais au moins il y a une ligne directrice un horizon d'attente générale qui est défini par le politique et qui, qui nous permet de, de discuter, tout le monde a insisté sur la nécessité de retravailler sur le continuum entre le lycée et la licence, c'est absolument fondamental, je vois à mon petit niveau, que les enseignants de l'université connaissait le bac dans son ancienne formule il siégeait dans dans les commissions, aujourd'hui ils sont dans l'incapacité, très souvent de comprendre ce qui se passe réellement au lycée et dans le bac, donc il faut absolument rapprocher les uns des autres et je crois qu'il y a d'abord un, un travail de formation des enseignants à faire sur ce qu'est l'université pour les hein et ce qui est le lycée pour pour les autres, je vais très vite sur les algorithmes locaux comme tout le monde est est déçu que que j'en ai pas parlé, ce que ce que tout le monde souhaite, Madame la Ministre, mais je crois que vous êtes d'accord c'est que il y ait une information sur les méthodes utilisées par par les jury pour trier préalablement dans des fichiers Excel, généralement c'est ça les dossiers des étudiants aujourd'hui ces données ne sont pas disponibles, il faut qu'elle le soit ex-hantée et je crois que c'est très important que dans les rapports qu'on a consulté ce que nous envoyer France France Université aujourd'hui, ces critères ne sont pas précisés, l'étudiant, le candidat pardon a besoin de savoir qu'est-ce que vos Manod de maths qu'est-ce que vous, et caetera, il y a une demande très forte que que je relaie ici sur le caractère qui doit être rendu le plus possible anonyme du lycée d'origine, on a le sentiment, les, les candidats ont le sentiment qu'ils sont aujourd'hui classés en fonction de leur lycée d'de d'origine, bien évidemment, c'est un billet, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à l'esprit, réplique hein de de l'université, je vais m'arrêter là, ce que j'ai déjà dépassé mon temps, merci monsieur le président. Merci, chers collègues, je vous remercie tous pour ce débat, et Madame la Ministre, pour ses réponses, mes chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance aura lieu le mardi 15 novembre à 14 heures 30 pour les explications de vote des groupes puis le scrutin public solennel sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 la séance est levée.